concerne les tests salivaires et les autotests dans les écoles. Cependant, il se pourrait bien que les autotests et les tests salivaires deviennent, dès la rentrée prochaine, le complément indispensable de la politique en faveur du vaccin, du vaccin, pour les plus de 12 ans et plus encore pour les enfants au-dessous de cet âge. Alors que le rythme de croisière de 300 000 tests par semaine, prévu initialement pour la mi-mars, a été atteint tardivement en fin d'année scolaire, fin d'année scolaire, des équipes enseignantes ont relevé de nombreux couacs dans la mise en oeuvre de cette stratégie de tests sur le terrain. Les délais entre la flambée des cas dans certaines écoles et l'arrivée des tests salivaires ont souvent été un peu longs.

Il semble donc urgent de préparer dès à présent les mesures sanitaires qui seront appliquées dans nos écoles à la rentrée, car elles seront un vecteur important de lutte contre la propagation du virus. Il semble aussi opportun de donner l'autorisation aux collectivités locales de lancer des campagnes massives de tests

de dépistage par test PCR sur prélèvement salivaire, plus de 4 millions de tests ont été proposés aux élèves et aux personnels travaillant dans les écoles et les établissements scolaires.

et des savoir-faire. C'est pourquoi il a droit à une éducation manuelle, qui est un levier puissant pour comprendre, apprendre, progresser et se construire. La main et le cerveau sont liés et travaillent ensemble. Nous sommes nés de cela, nous avons évolué grâce à cette synergie, et ce depuis l'aube de l'humanité. Alors que notre société est de plus en plus informatisée, numérisée, dématérialisée, alors que nous avons tant besoin de prise directe avec la réalité, alors que nos enfants grandissent beaucoup trop devant les écrans, pourquoi les priver de ce ressort magnifique de connexion avec le réel, de ce chemin de facilité vers la connaissance ? Faire avec ses mains permet d'aider à acquérir toutes les notions et à les consolider, y compris les notions les plus abstraites et les plus intellectuelles. Sinon comment un élève qui n'a pas la chance d'avoir des parents artisans ou bricoleurs, qui n'a donc pas vu, senti, vécu ni essayé le travail manuel et qui n'a plus goût à l'école peut-il savoir qu'il est fait pour travailler manuellement, qu'il va aimer cela et qu'il sera heureux heureux d'embrasser une profession manuelle, laquelle lui permettra de se réaliser ? Nous sommes nombreux à avoir grandi en suivant des cours d'éducation manuelle. De tels cours manquent cruellement aujourd'hui. Si tous les enfants pouvaient, durant leur scolarité, s'essayer à la menuiserie, à la couture, à la poterie, à la cuisine, au tricot, à la vannerie et à mille autres choses, ils pourraient s'orienter en connaissance de cause. Ils seraient alors certains qu'ils peuvent trouver là les moyens de s'accomplir. La pandémie a été riche d'enseignement : l'éducation manuelle aurait été d'un grand secours, ne serait-ce que pour faire un masque. Imaginez comment les enfants auraient pu participer, s'investir dans l'élan de solidarité nationale et dans cette situation si difficile à vivre en tant qu'acteurs impliqués, être reconnus et faire partie de ceux qui ne sont pas restés uniquement sidérés ! Lors de la discussion du projet de loi pour une école de la confiance,

comprise comme l'ensemble des « activités d'investigation, de conception, de modélisation et de réalisation » est présente et a vocation à être renforcée, de la maternelle au lycée. Cette omniprésence permettra aux élèves d'acquérir des compétences encore plus larges

l'action du Gouvernement en faveur de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, visible ou invisible, n'est pas très claire. La Fédération française du sport adapté organisera à Vichy en 2023 les, accueillant ainsi près de 1 000 athlètes du monde entier dans dix différentes disciplines sportives. En 2024, Paris accueillera les jeux Paralympiques, qui rassembleront, quant à eux, plus de 10 000 athlètes pour près de 330 épreuves. Les sont un événement phare et une chance pour les sportifs de haut niveau ayant une déficience intellectuelle.

Malgré un réel engagement pour Paris 2024 et les jeux Paralympiques, il est regrettable qu'aucune action de promotion ou de soutien n'ait été prise pour le moment par le Gouvernement pour cet événement majeur qui se déroulera à quelques mois des jeux Paralympiques.

qui ne pouvait pas être parmi vous ce matin. Portée par la Fédération française du sport adapté, la candidature de Vichy pour l'accueil de la plus grande compétition internationale de sport adapté avait été dévoilée des 2019 par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et par Sandrine Chaix, conseillère spéciale régionale au handicap.

Les 2023 sont inscrits au calendrier des grands événements paralympiques internationaux par la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, et sont soutenus à hauteur de 700 000 euros pour un budget de 3,256 millions d'euros, soit 21 % de taux de soutien. L'Agence nationale du sport accompagne également la Fédération française du sport adapté et tous ses sportifs de haut niveau au travers d'un contrat de performance, à hauteur de 900 000 euros en 2021.

au travers de la Fédération, que ce soit pour les trois sports paralympiques- athlétisme, natation, tennis de table -ou pour les sports non paralympiques reconnus de très haut niveau. J'espère, monsieur le sénateur, que ces éléments d'information ont pleinement répondu à votre question. La parole

souligné l'engagement fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec son président Laurent Wauquiez et sa vice-présidente Sandrine Chaix, qui se mobilisent fortement pour l'organisation de l'édition 2023. Vous avez évoqué l'édition 2019, et

telles que l'Ossau-Iraty au système du Nutri-score. Ce fromage au lait de brebis, fabriqué dans les Pyrénées-Atlantiques, est classé en appellation d'origine contrôlée (AOC) depuis 1980 et en appellation d'origine protégée (AOP) depuis 1996. Il s'agit d'un produit traditionnel, de grande qualité, tant par sa fabrication-du lait cru non chauffé -que par le mode d'élevage de la filière ovine concernée : le pâturage en estives basco-béarnaises. Or cette spécialité est aujourd'hui confrontée à un déficit d'image en raison du dispositif Nutri-score qui lui est appliqué. En effet, elle est classée D dans cette grille, alors que des produits industriels transformés se voient paradoxalement attribuer des notes bien meilleures. À un moment où le consommateur souhaite légitimement être informé des produits qu'il va trouver dans son assiette, il est paradoxal que le Nutri-score, qui limite l'information à la simple composition nutritionnelle, devienne prédominant. Il convient de le rappeler, le cahier des charges des AOC et AOP est très strict et les modes de fabrication ainsi que la composition des produits ne peuvent pas être modifiés, ce qui ne permet pas d'adapter leur composition pour répondre aux exigences du Nutri-score. De plus, Santé publique France envisage d'interdire la publicité des aliments notés D et E pour préserver les enfants et adolescents du marketing publicitaire, ce qui entraînera l'impossibilité d'assurer la promotion de tels produits sous indication géographique. Cette situation me semble aller à l'encontre

serait-il envisageable de ne pas soumettre les productions traditionnelles au système du Nutri-score, celui-ci paraissant inadapté dans ces cas-là ? La parole

pour les consommateurs en termes de qualité, de savoir-faire, de protection de l'environnement, d'origine et de terroir, alors que le Nutri-score les informe sur la qualité nutritionnelle des produits transformés et permet donc de les comparer. Si les fromages sont

en lien avec le ministère de la santé, que le comité scientifique institué au niveau européen se saisisse de la question des fromages, afin de mieux traduire la corrélation entre les teneurs en protéines et en calcium des fromages. Quoi qu'il en soit, cela ne doit pas pour autant exclure ces produits

et soutenir. Nous pensons qu'il vaut mieux nous pencher sur les spécificités nutritionnelles des produits sous AOP. Ainsi, sept pays sont désormais engagés dans cette démarche : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Un comité composé d'experts scientifiques, réuni pour la première fois le 12 février dernier, aura pour mission d'évaluer la pertinence

En effet, dans les Hauts-de-France, on joue énormément « à pigeons », on enchaîne les courses. Les colombiers cultivent le bien-être animal, la convivialité et la compétition sportive. Si j'ai décidé d'introduire mon propos de cette façon, c'est pour mettre en exergue un aspect important de ce sport : le lien social. C'est un lien fort et unique qui lie entre eux les colombophiles non seulement européens, mais aussi britanniques. comme chacun sait, le Brexit est arrivé et avec lui son cortège de complications. Les pigeons voyageurs en provenance du Royaume-Uni bénéficiaient, jusqu'alors, autorisation d'introduction sur le territoire français. Dorénavant, ils ne peuvent plus être transportés aussi facilement et le lien qui unit les passionnés des deux côtés de la Manche en pâtit. C'est le règlement européen 2020/692 qui régit dorénavant les importations d'oiseaux captifs, dont les pigeons voyageurs. Ce dernier impose une quarantaine de trente jours, mettant en difficulté la tenue des compétitions colombophiles. Je sais que cette problématique a été prise en compte et que le texte européen est en cours de modification. En attendant, les pigeons voyageurs sont naturellement soumis aux dispositions nationales. À ce jour, les postes de contrôle frontaliers des Hauts-de-France- Dunkerque, Calais port et Calais tunnel -ne sont pas en mesure d'assurer le contrôle à l'importation de ces animaux. j'aimerais donc vous poser deux questions. Pouvez-vous m'informer, d'une part, de l'état d'avancement de la modification du texte européen ? Acceptez-vous, d'autre part, de prendre des dispositions pour permettre aux postes

Vous l'avez dit, des travaux sont actuellement engagés par la Commission européenne : ils devraient conduire à la parution d'un acte délégué modificatif du règlement, spécifiquement dédié aux nouvelles modalités d'importation en provenance des pays tiers. La date de parution de cet acte

les importations sont actuellement possibles sous couvert du respect des dispositions nationales fixées par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2002. Ce texte impose notamment que tous les animaux vivants en provenance des pays tiers soient soumis aux fameux contrôles vétérinaires d'introduction dans un poste de contrôle frontalier. À ce jour, et cela répond à votre seconde question, à votre seconde question, seuls les postes de contrôle frontalier de Caen-Ouistreham, de Cherbourg et de Saint-Malo sont désignés et disposent des infrastructures adaptées pour le contrôle de ces animaux sur la façade Manche. Vous l'avez dit, ce n'est pas tenable Les demandes d'extension du champ de désignation d'autres postes de contrôle frontaliers relèvent non pas de la compétence du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, mais de celle des gestionnaires des points d'entrée- ports et tunnels -au regard de leur appréciation de l'opportunité d'investir dans des infrastructures nécessaires, considérant les flux attendus. Aussi, si ces derniers l'estiment opportun, ils peuvent présenter un dossier de désignation, qui sera bien évidemment étudié par les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation avec attention, en particulier par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, puis transmis à la Commission européenne afin de recueillir son accord. Monsieur le sénateur, je tiens à vous assurer que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est attaché comme vous au lien social que cette

de rendre obligatoire un stage en PME pour les étudiants des grandes écoles, comme l'École nationale d'administration (ÉNA), l'École polytechnique ou encore l'École nationale supérieure des Mines de Paris. En effet, bien que la situation sanitaire actuelle occupe une grande partie des actions menées par le Gouvernement, il est essentiel de ne pas mettre de côté des initiatives qui pourraient aider les entreprises, notamment les plus petites, PME et les très petites entreprises (TPE). En 2015, 63 % des salariés étaient employés dans une PME, mais ces entreprises embauchent beaucoup moins de jeunes diplômés que les grandes sociétés. Or cela leur porte préjudice, car de nombreuses études montrent l'importance de ces profils pour le développement mais aussi pour le dynamisme D'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, se sont saisis du problème et ont mis en place des programmes spécifiques associant grandes universités et PME et facilitant les stages. En Allemagne, le niveau moyen d'encadrement des entreprises est bien meilleur que celui des PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, notamment parce que les jeunes diplômés s'y orientent naturellement à la sortie de leurs études. Il paraît donc opportun de faire découvrir aux futurs grands décideurs ce qui fait notre richesse économique. Trop souvent, les étudiants des grandes écoles intègrent directement de grands établissements, privés ou publics, ce qui ne les confronte pas à la diversité économique de notre pays et de nos territoires. Nos dirigeants sont par ailleurs très demandeurs de ce type d'initiative et la Banque publique d'investissement, Bpifrance, y a déjà travaillé. C'est une volonté forte exprimée par les réseaux de petites et moyennes entreprises. Il me semble donc primordial d'instaurer, de manière systématique, au moins un stage dans une petite entreprise dans le cursus des étudiants de nos grandes écoles françaises. vouloir m'indiquer, madame la ministre, ce que le Gouvernement compte faire sur ce sujet.

de leurs étudiants. Ainsi, à l'ÉNA, les élèves suivent un stage de sept mois en préfecture ou en collectivité territoriale, au cours duquel ils effectuent une « mission entreprise » de deux mois,

dans le cadre de l'Institut national du service public, qui sera créé au 1 janvier 2022, ces stages en entreprise seront pérennisés et l'ouverture des élèves sur le secteur privé sera renforcée par la création d'un tronc commun à toutes les écoles de service public. Toujours dans la même dynamique, l'Institut national des études territoriales prévoit un stage d'ouverture de quatre semaines pouvant s'effectuer dans le secteur privé. Le Centre national de la fonction

Ainsi, les élèves ingénieurs de l'École supérieure des Mines ParisTech passent au minimum douze mois en entreprise sur les trois années de formation. Le Gouvernement est par ailleurs attaché au renforcement des liens entre l'ensemble des étudiants et le tissu des PME de nos territoires. Les volontariats territoriaux en entreprise permettent, par exemple, à des étudiants du supérieur d'avoir des expériences en PME industrielle, avec des soutiens financiers. L'apprentissage est également un levier puissant d'accueil d'étudiants dans des PME.

et de l'innovation. Madame la ministre, j'appelle votre attention sur la licence professionnelle consacrée au bois et à l'ameublement du lycée Charles-de-Gaulle de Chaumont, en Haute-Marne. Cette licence professionnelle consacrée au bois et à l'ameublement, avec option « création et du cadre de vie » ne devait plus être dispensée dans le lycée, à partir de la rentrée 2021. Cette décision a provoqué une grande incompréhension dans le département, alors que cette formation est dispensée depuis huit ans et que, l'année dernière, pas moins de 70 candidatures ont été reçues pour seulement 15 places. Fort heureusement, cette décision ministérielle a été annulée après la mobilisation de nombreux acteurs contre cette fermeture, et je m'en réjouis. Ce que je regrette, en revanche, c'est le manque de concertation entre le Gouvernement, l'université et ses enseignants, ainsi que les élus locaux et les chambres consulaires. Si cette décision avait été justifiée, elle aurait été acceptée, probablement. Dans ce cas précis, elle ne l'était pas, bien au contraire. La filière bois a un réel avenir sur notre territoire, puisque notre département possède désormais le premier parc national des forêts de plaines et de nombreux atouts dans ce domaine. domaine. Des efforts ont été réalisés pour dynamiser notre territoire et offrir des formations post-bac aux jeunes du territoire, en adéquation avec notre environnement et nos projets économiques et touristiques. Par conséquent,

formations pourvoyeuses d'emplois. Par conséquent, que compte faire le Gouvernement pour que les formations en lien avec la filière bois perdurent dans le département de la Haute-Marne et que les jeunes puissent ensuite y travailler et y vivre ?

Néanmoins, la formation proposée n'était pas conforme à la réglementation applicable aux licences professionnelles, avec notamment un nombre trop faible d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants universitaires au sein de l'équipe pédagogique. L'accréditation avait par conséquent été donnée pour trois ans et assortie d'une demande de réexamen à mi-parcours ; ces trois années devaient permettre à l'université de se mettre en conformité avec la réglementation, en garantissant le caractère universitaire de la formation. L'université de Reims Champagne-Ardenne a transmis, en octobre 2020, un dossier de demande de prolongation de l'accréditation pour cette licence. Cette demande a été instruite par le collège des conseillers scientifiques et pédagogiques de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle qui a sollicité des compléments d'information auprès de l'université, notamment des données chiffrées portant sur l'insertion professionnelle et sur la composition de l'équipe pédagogique. L'université a répondu à cette demande, mais la réponse apportée a été jugée insatisfaisante sur les deux aspects cruciaux de la formation professionnalisante

tant sur l'implication de l'université que sur les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque année, environ 2 000 licences professionnelles sont accréditées par le ministre, ce qui représente plus de 52 000 étudiants. Il s'agit d'un diplôme phare de l'université,

À l'inverse, depuis plusieurs années, on observe une augmentation importante du nombre de places en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). Cette évolution s'explique par une volonté d'accompagner les enfants dans les différents lieux dans lesquels ils évoluent quotidiennement et de développer l'école inclusive, démarche qui est à saluer. Toutefois, l'augmentation du nombre de places en Sessad se fait au détriment du nombre de places en ITEP et en IME. Or nombre d'enfants en situation de handicap ne peuvent être accompagnés dans ce format externalisé et doivent être suivis dans des établissements spécifiques et équipés pour les accueillir.

du nombre de places entre, d'un côté, les ITEP et les IME, et, de l'autre, les Sessad, afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap.

Cette transformation conduit à réviser les équilibres de répartition de places entre solutions d'hébergement en structure spécialisée et services d'accompagnement à domicile et en milieu ordinaire,

Aujourd'hui, nous créons des unités d'enseignement spécialisé- les classes adaptées pour les autistes et les classes externalisées -afin de mettre en oeuvre cette coopération si indispensable. Nous créons aussi des formations

Face à ce manque de place, les enfants étaient redirigés vers les unités localisées pour l'inclusion scolaire, les fameuses ULIS, en lien avec l'éducation nationale. Parfois,

(SDREA) régule l'accès des exploitants au foncier agricole en fonction des enjeux nationaux et locaux. Ce schéma, encadré par les articles L. 331-1, 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soumet certaines opérations de mise en valeur des terres- installation, agrandissement ou réunion d'exploitations -à autorisation préalable. Il est particulièrement utilisé pour permettre aux petites structures d'être privilégiées par rapport aux grandes exploitations, dans l'obtention de l'autorisation d'acquérir et d'exploiter les terres agricoles libérées. Il permet de lutter contre la concentration excessive des terres et de consolider les petites exploitations. Il paraît néanmoins que, même si le schéma permet aux agriculteurs français d'être mis en concurrence dans des conditions justes et équitables, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'agriculteurs étrangers frontaliers, qui sont nombreux, notamment dans la région Grand Est. Alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français et que l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive sont prises en compte, seules les terres exploitées par un agriculteur étranger en France sont comptabilisées et soumises au contrôle administratif du préfet. Les agriculteurs étrangers sont donc favorisés si la majeure partie de leur exploitation est située à l'étranger. Il en résulte une distorsion flagrante de concurrence puisque les agriculteurs français ont plus de difficultés à obtenir l'autorisation d'exploiter de nouvelles terres agricoles. Cette situation ne peut se résoudre uniquement à l'échelon national. Même si le code rural exige de prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, le Gouvernement français doit agir à l'échelon européen pour faire respecter l'équité et la libre concurrence entre tous les agriculteurs.

Si tout agriculteur, quelle que soit sa nationalité, doit respecter les dispositions du contrôle des structures sur notre territoire, la loi française est soumise au principe de territorialité. Les terres exploitées à l'étranger ne sont ainsi pas soumises au contrôle administratif du préfet. Mme Belrhiti défend l'idée d'une action à l'échelon européen pour résoudre ces difficultés. L'Union européenne a marqué son intérêt, au cours des dernières années, pour les questions relatives à la régulation du foncier agricole

de la Commission sur l'acquisition de terres agricoles et le droit de l'Union européenne. La réflexion mérite d'être poursuivie. Pour autant, l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose : « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. Les règles régissant l'utilisation des terres agricoles relèvent ainsi de la compétence des États membres. La possibilité de tendre vers un cadre de réglementation harmonisé à l'échelon européen me semble donc très hypothétique au regard de la complexité du sujet et de contextes différents, y compris entre pays frontaliers. Si les circonstances locales le justifient, des solutions peuvent être toutefois trouvées dans la coopération transfrontalière. Je peux ainsi citer les travaux menés dans le cadre de la conférence transjurassienne : à cette occasion, les autorités françaises et suisses ont mis en place une commission technique de conciliation foncière, qui permet de coordonner la régulation du foncier entre les deux pays. Cette commission a permis de mettre en place un protocole de suivi des exploitants suisses en France relevant d'une collaboration entre l'administration française, dans les départements du Doubs et du Territoire de Belfort,

depuis maintenant deux ans, je me mobilise pour des familles demeurant dans le département dont je suis élue, le Pas-de-Calais, plus particulièrement dans la commune de Leforest, victime de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de 2018. En août 2019, le maire de cette commune a été contraint de prendre un arrêté de péril imminent relatif à certaines habitations, forçant ainsi des familles à quitter leur domicile. En effet, ces logements étant construits sur une zone argileuse, une zone argileuse, qui se gonfle ou se rétracte au gré des épisodes météorologiques, d'importantes fissures sont apparues sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments, à la suite de l'épisode de sécheresse de 2017 ; depuis lors, elles ne cessent de s'étendre. les familles continuent de payer des traites pour les maisons qu'elles ne peuvent plus habiter et doivent, en outre, s'acquitter des loyers des logements dans lesquels elles ont dû évacuer. Les difficultés semblaient inextricables jusqu'à une excellente nouvelle, datant de samedi dernier : la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des communes supplémentaires touchées par la sécheresse de 2018, dont Leforest. Je me réjouis de cette annonce, qui récompense la mobilisation des élus, des associations et de la commission interparlementaire créée à cette occasion, pour que justice soit rendue à ces communes touchées.

La toute récente reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Leforest doit maintenant permettre l'indispensable indemnisation de ces familles.

Il s'agit d'assurer que ce type de dégâts ne se reproduise pas pour les constructions à venir. À plus court terme, afin de remédier à certaines situations d'urgence liées à la sécheresse de 2018, la loi de finances pour 2020 a prévu la mise en place exceptionnelle, à hauteur de 10 millions d'euros, d'un dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par la sécheresse de 2018. Ce fonds, forcément limité, doit en priorité aider les ménages qui se trouvent dans les situations les plus difficiles. Ainsi, sont éligibles uniquement les travaux lourds et coûteux, qui nécessitent une intervention sur la structure ou les fondations. Il a également paru nécessaire de cibler prioritairement les propriétaires aux revenus modestes, qui n'auraient pu réaliser de tels travaux sans cette aide. Cela étant, comme vous le soulignez, la typologie des demandes reçues depuis la mise en place de ce fonds a conduit à étudier son ouverture à des ménages aux revenus intermédiaires.

Inspection générale de l'administration et Conseil général de l'environnement et du développement durable -, qui ont remis leur diagnostic et leurs propositions en mai dernier. Sur le fondement de ce travail, certaines dispositions législatives nouvelles pourraient être introduites, la proposition de loi du député Stéphane Baudu portant sur ce sujet.

par la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, déterminant la qualité de travailleur frontalier, au bassin d'emploi de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Cet établissement a été institué sous la forme d'un par la convention du 26 avril 2010, signée par la France, l'Espagne et la Généralité de Catalogne. Cette convention a été suivie par la ratification de l'accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière entre la République française et le Royaume d'Espagne, autorisée par le Parlement, au travers de La vocation première de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne, situé côté espagnol, dans la commune de Puigcerdà, est de fournir des soins médicaux aux habitants du plateau de Cerdagne, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole. Il s'agit d'une population d'environ 30 000 personnes, qui n'avaient pas d'accès facile aux soins, leur région montagneuse étant enclavée. De façon logique, le bassin d'emploi de l'hôpital correspond à sa zone de compétence plateau de Cerdagne est un peu plus étendu que la zone frontalière prévue par la convention fiscale franco-espagnole. Le rayon prévu par cette convention n'est que de 20 kilomètres de part et d'autre de la frontière, mais il s'avère manifestement insuffisant, car nombre d'employés de l'hôpital habitent au-delà, quelquefois même

pour définir les déplacements transfrontaliers lors des derniers confinements liés à la pandémie de la covid-19. Je souhaite donc savoir, madame la ministre, si le Gouvernement envisage de modifier la convention fiscale franco-espagnole afin d'élargir cette zone transfrontalière et, dans l'affirmative, dans quel délai.

frontalier spécifique. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises, puis intégré dans sa forme actuelle dans la convention, actuellement en vigueur, du 10 octobre 1995. Le point 12 du protocole de la convention garantit aux travailleurs frontaliers d'être imposés sur leurs revenus d'activité dans l'État dont ils sont résidents. Conformément à l'article 2 de l'accord complémentaire entre la France et l'Espagne relatif aux travailleurs frontaliers, le statut de frontalier est reconnu aux travailleurs résidant dans une liste limitative de communes situées à une distance de 20 kilomètres au plus de la frontière espagnole. Il est précisé que ce régime est tout à fait comparable, sous cet aspect, à celui qui a été conclu avec les autres pays frontaliers, la Belgique et l'Allemagne par exemple. La question des travailleurs frontaliers, et plus particulièrement la révision du régime prévu, peut difficilement être envisagée sous le seul angle des besoins exprimés par les travailleurs de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. En effet, une extension à 30 kilomètres de la zone frontalière aurait, par construction, des conséquences plus larges et générales. La modification de ces règles devrait nécessairement passer par un accord bilatéral, ce qui suppose un accord de nos partenaires espagnols et une révision de la convention,

C'est pourquoi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'extension de la zone transfrontalière que vous évoquez dans votre question, et dont la pertinence est pleinement reconnue, n'est pas envisagée à ce jour. La parole est à M. François Calvet, pour la réplique.

qui, certainement par nécessité, continue à appliquer les mêmes méthodes que dans l'Hexagone, alors que la situation de la Guyane est toute particulière et, surtout, très différente.

il faudrait y ajouter les enquêtes de terrain, les données sur la consommation d'eau et d'électricité et le volume des déchets si l'on veut parvenir à une fiabilité en matière de recensement. Pour illustrer mes propos, et à titre d'exemple, alors que la croissance annuelle moyenne sur les dix dernières années est de 2,6 %, l'Insee n'a pas hésité à publier une croissance de la population négative pour 2020, à-0,26 % ! C'est une première. Qui peut le croire, à part l'Insee

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Georges Patient, votre question m'invite à vous répondre en deux temps. En ce qui concerne la croissance de la population guyanaise en 2020, les populations légales des communes de Guyane intègrent, depuis le début de l'année 2020, une rénovation dans la méthode de recensement des zones d'orpaillage clandestines. Cette rénovation vise à en améliorer la précision et à assurer l'égalité de traitement des communes guyanaises entre elles et avec le reste du territoire français, afin de fiabiliser les chiffres utiles pour l'édiction des dispositions réglementaires qui en découlent. Désormais, la collecte dans ces zones fait l'objet de contrôles qualité renforcés de l'Insee. Lorsque, pour des raisons de sécurité, la collecte sur le terrain n'est pas possible, la population de ces zones est mise à jour la préfecture de Guyane, à partir des données de l'Observatoire de l'activité minière. Ce n'était pas le cas auparavant, ce qui conduisait à une surestimation du nombre de personnes résidant dans les zones d'orpaillage. L'évolution des populations légales des communes guyanaises entre 2019 et 2020 traduit l'ajustement opéré pour corriger cette surestimation. Elle ne doit pas être confondue avec l'évolution démographique de la population résidant sur ces territoires, qui s'est poursuivie selon la même dynamique. En ce qui concerne le report des opérations de recensement sur le terrain en 2021 et l'actualisation des populations légales au 1 janvier 2022, l'Insee a engagé des travaux méthodologiques pour disposer d'estimations fiables, en l'absence de collecte sur le terrain. Les premiers résultats ont fait l'objet d'une présentation devant la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population le 13 avril dernier. La qualité des estimations de populations obtenues est pleinement satisfaisante et lève les craintes que l'actualisation des populations légales, dans le contexte d'un report de l'enquête annuelle de recensement, a pu susciter.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

une taxe sur la première cession d'un terrain rendu constructible s'applique indifféremment de la qualité du cédant, qu'il soit une personne physique ou morale. À ce titre, une commune doit acquitter la taxe dès lors qu'elle réalise une plus-value sur la vente d'un terrain qu'elle aura rendu constructible. Or la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Ainsi, l'ensemble des travaux inhérents à la viabilisation du ou des terrains, les études d'urbanisme et autres frais engagés pour la réalisation d'un lotissement, par exemple, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value. L'augmentation du prix de vente du terrain, qui permettrait d'imputer indirectement la taxe afin que la commune ne réalise pas une opération déficitaire, ne constitue pas une solution de pour de nombreuses communes rurales qui souhaitent développer leur territoire et qui manquent de logements pour répondre aux besoins des salariés des entreprises environnantes. Cela est d'autant plus irréaliste dans le cas de logements sociaux. nous avons eus hier soir sur l'urbanisme et le logement attestent des difficultés et des freins rencontrés par de nombreuses communes, lesquels s'ajoutent au désintérêt des opérateurs. C'est pourquoi, madame la ministre, je vous demande s'il est envisageable de revoir la méthode de calcul de la taxe prévue à l'article 1605 du CGI. La parole Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Annick Billon, comme vous l'indiquez, la taxe prévue à l'article 1605 du code général des impôts s'applique aux cessions de terrains nus rendus constructibles. Les cessions de terrains nus faisant l'objet d'un lotissement sont soumises à cette taxe, qui s'applique quelle que soit la qualité du cédant- personne physique ou personne morale de droit privé ou de droit public -et sans égard pour le régime fiscal de La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession diminué du prix d'acquisition. Ce prix d'acquisition correspond au prix stipulé dans l'acte ou, à défaut, à la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant. Le prix de cession est calculé d'après les mêmes règles que celles qui sont applicables en matière d'imposition des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu. Ainsi, ce prix de cession peut être réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et de certains frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Les frais engagés pour la cession peuvent donc être déduits, sous réserve qu'ils soient explicitement listés par le code général des impôts. Par exemple, peuvent être déduits les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire, les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession, les honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable au permis de construire ou encore les frais de mainlevée d'hypothèque. En revanche, ce droit à déduction ne s'étend pas, comme à l'impôt sur le revenu, à des dépenses telles que les frais de viabilisation des terrains cédés, qui ne sont pas directement liés à la cession. Par ailleurs, il convient de relativiser les inconvénients de ces règles de calcul pour les collectivités. Tout d'abord, cette taxe ne s'applique que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, c'est-à-dire pour les plus-values substantielles. Ensuite, les règles de calcul de la taxe assurent que le montant dû ne soit pas trop élevé, un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible, avec des taux modérés. Il est difficilement envisageable de modifier ces règles uniquement pour les collectivités, qui ne constituent que des redevables de la taxe parmi d'autres, au risque de créer une rupture d'égalité devant l'impôt. autoriser la déduction des frais de viabilisation serait incohérent avec les objectifs de cette taxe, qui, je vous le rappelle, a pour effet de freiner la transformation de terres agricoles en terrains à bâtir. Son produit est ainsi affecté à un fonds qui finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture.

et de la relance. Madame la ministre, en juin 2020, la papeterie normande Chapelle Darblay, unique entreprise à fabriquer du papier 100 % recyclé en France, fermait, malgré sa rentabilité, en raison, selon son propriétaire finlandais UPM, d'un manque de compétitivité et du déclin structurel du papier journal. Cette usine, fleuron de l'économie circulaire en activité depuis près d'un siècle, pouvait absorber jusqu'à 480 000 tonnes de papier à recycler par an, soit le résultat du tri de 24 millions d'habitants. Dans l'espoir d'une reprise, elle n'a pas été démantelée. Depuis sa fermeture, ses machines et sa chaudière biomasse sont dormantes, mais restent utilisables. Les repreneurs avaient jusqu'au 30 juin 2021 pour se signaler. Or, le 2 juillet, le propriétaire de l'usine a présenté, dans le cadre d'un comité social et économique exceptionnel, une offre de rachat pour le moins étonnante, puisqu'il s'agit d'une transformation du site en une unité de production d'hydrogène. Cette offre, issue d'un acteur qui se positionne partout en France, reprendrait seulement partiellement les pièces des machines du site. Elle n'implique ni fret maritime ni fret fluvial et prévoit seulement 70 emplois- pour rappel, ce sont 230 personnes qui ont été licenciées en juin 2020, lors de la fermeture du site. Référence en matière de transition écologique, Chapelle Darblay représente un important savoir-faire en matière de recyclage, secteur dont l'avenir ne fait aucun doute. Dans une lettre d'intention, Veolia, géant du traitement de l'eau et des déchets, a présenté, avec deux partenaires, un projet de reprise sérieux et cohérent, qui permettrait de prolonger son activité papetière. Ce groupe a besoin de trois mois pour finaliser ce projet et le transformer en offre concrète. Je me réjouis, dans ce contexte, que, grâce à la mobilisation des salariés de l'usine, la décision finale ait été retardée au mois de septembre Compte tenu de l'intérêt de ce projet, qui préserve les compétences de Chapelle Darblay, et de l'engagement pris par le Gouvernement en matière de transition écologique, je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir intervenir auprès du propriétaire de ce site pour en assurer la sauvegarde à tous points de vue et de m'indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre en ce sens.

Celle-ci travaille activement à la reconversion du site emblématique de Chapelle Darblay, en instance de cession par son propriétaire, le groupe finlandais UPM. Je ne vous apprends rien : ce site a dû fermer il y a un an faute de repreneur, dans un contexte sanitaire défavorable. Le Gouvernement a oeuvré pour favoriser une reprise, aux côtés des représentants du personnel, dont nous saluons l'implication décisive. L'État a engagé une troisième prospection de septembre 2020, Business France, aux côtés de la région Normandie. En parallèle, ma collègue a confié une mission au Conseil général de l'économie pour déterminer des pistes de reconversion durable pour Chapelle Darblay. Le marché du papier journal étant en forte décroissance, la pérennité de l'emploi et de l'activité industrielle exigeait de nouvelles perspectives. De plus, des pistes de valorisation des actifs présents sur le site, en particulier de la chaudière de biomasse et de la station d'épuration, ont été recherchées. Le Gouvernement et les services de l'État sont en contact direct avec plusieurs acteurs industriels. Enfin, la convention de revitalisation conclue entre l'État et UPM prévoit le versement de 500 000 euros par UPM, attribués au projet de reprise du site. Comme vous le savez également, à quelques kilomètres de Chapelle Darblay, une autre papeterie produisant du papier d'impression et comptant 180 emplois, Alizay, se trouvait en grande difficulté. Nous avons pu garantir la reprise de ces deux sites papetiers normands. Pour chacun d'eux, nous avons une solution d'avenir. Alizay est reprise par le cartonnier VPK et deviendra un grand pôle de recyclage, avec la production de papier carton pour emballage et la construction d'une usine de recyclage de papiers. Ces productions bénéficieront de l'énergie verte produite par une chaudière biomasse. À Chapelle Darblay, l'offre de reprise que vous avez mentionnée est portée par deux groupes, Samfi et Paprec, dont les activités sont complémentaires. 70 emplois seront créés à court terme par l'entreprise Paprec, spécialiste du recyclage et de la valorisation des déchets, 140 emplois supplémentaires seront créés par le groupe Samfi et sa filiale H2V, pour la production d'hydrogène. Nous parlons donc de 210 emplois au total. Quant à l'entreprise Veolia, présente dans la procédure depuis plus d'un an, elle n'a pas souhaité déposer d'offre ferme pour la reprise de Chapelle Darblay. La lettre d'intention transmise à quelques jours de la fin de la procédure n'a pas suffi à assurer un caractère sérieux. Nos objectifs sont néanmoins remplis : la filière du recyclage en Normandie, l'activité industrielle à Chapelle Darblay et Alizay et 400 emplois seront maintenus et assurés. La parole

ce qui nous convient. Nous souhaitons que le Gouvernement s'engage fortement en faveur d'une reprise par Veolia, en accompagnant ce projet dans tous les domaines qui puissent le faire aboutir. La parole est à M. Joël Labbé, auteur

recherche médicale (Inserm) rappelle et alimente ce triste constat : l'exposition aux pesticides a bien un effet sur la santé- en premier lieu, sur celle des utilisateurs, mais aussi sur celle des riverains. accessible à tous- la loi Égalim -, malgré une injonction du Conseil d'État de 2019 à revoir la réglementation sur les pesticides, la réponse apportée est toujours plus que décevante. Elle consiste, en effet, à la mise en place de chartes départementales, supposées définir des règles de « bon voisinage », mais dont la fonction essentielle, sur le terrain, est de permettre de déroger aux distances d'épandage fixées par les textes, pourtant très réduites. Sources majeures de tension à l'échelon local, ces chartes ont été attaquées et, en mars dernier, le Conseil constitutionnel les a jugées non conformes, estimant que la procédure de participation prévue pour leur élaboration ne respectait pas la Charte de l'environnement. Pas plus tard qu'hier, dans le cadre d'un nouveau recours, le rapporteur public, présentant ses conclusions, appelait le Conseil d'État à annuler les textes encadrant l'épandage des pesticides,

Le Gouvernement vient pourtant- au coeur du mois de juillet -d'inviter les préfets à mettre en consultation de nouvelles chartes, sans attendre la décision du Conseil d'État, prévue d'ici à quelques semaines. Ce passage en force est, pour nous, inacceptable. est, pour nous, inacceptable. Aussi, le Gouvernement prévoit-il de sortir de l'inaction sur ce sujet et de mettre en place de nouveaux textes qui soient réellement protecteurs

inconstitutionnelles les dispositions relatives à la mise en consultation des chartes d'engagements prévues par le code rural. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a relevé que la procédure particulière de concertation introduite dans le code rural

conformément aux dispositions du code de l'environnement doivent faire l'objet d'une consultation adaptée, donc de nouvelles discussions. Il me semble important de préciser que cette décision ne remet pas en cause les chartes, qui ont pour objet de formaliser les engagements des acteurs sur un territoire. C'est la manière dont elles ont été concertées, avec les parties prenantes, qui n'est pas conforme aux attendus du droit. Il convient également de rappeler que l'adaptation des distances de sécurité repose sur une série de mesures apportant des garanties en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et s'est rapidement mis en capacité de se conformer à cette décision. Un recensement des modalités précises de mise en consultation publique des chartes a ainsi été effectué. Monsieur le sénateur, je vous confirme l'ambition du Gouvernement de préserver la démarche vertueuse que constituent les chartes élaborées dans les départements. Celles-ci favorisent le dialogue entre les parties prenantes, dans l'intérêt de tous. je vous remercie en effet, de pesticides cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le ministre met en avant le label Haute Valeur environnementale (HVE), mais ce dernier permet de poursuivre l'utilisation de ces substances, particulièrement toxiques. On se rend compte que le Gouvernement aide à ce que l'on appelle « la modernisation de l'agriculture », en baissant les aides à l'agriculture qui n'utilisent pas ces produits. Nous espérons que les choses évolueront dans le bon sens

Ce petit bourg a su mettre en oeuvre, avec efficacité, une politique de développement qui porte ses fruits et il veut compléter son offre de services en créant un pôle santé. Il a déjà réussi à installer un cabinet d'infirmiers, de kinésithérapeutes et des discussions sont en cours en vue de l'installation d'un médecin. Mais, alors qu'un pharmacien est prêt à rejoindre ce pôle santé, l'autorisation d'ouverture d'une officine lui a été refusée. Dans sa réponse à ma question, la ministre avait ouvert une perspective d'assouplissement des critères, au travers de l'ordonnance du 3 janvier 2018.

Comment peut-on empêcher des professionnels de santé de s'installer dans des territoires ruraux, alors même que ces territoires doivent relever le défi de leur attractivité et d'une offre de soins qui s'est considérablement dégradée ? Madame la ministre,

dans le cas présent, en autorisant l'implantation d'une pharmacie dans la commune de Vézac ? La parole

La France est plurielle. Elle fait d'ailleurs une richesse de la diversité de ses territoires. Mais il nous faut prendre en compte cette diversité pour adapter les politiques publiques en conséquence et répondre à l'aspiration légitime de nos concitoyens à l'égalité dans l'accès aux soins et aux traitements.

de manière satisfaisante. Ainsi, les transferts d'officines dans ces territoires seront facilités et pourront se traduire par une installation, à proximité, par exemple, d'une maison de santé pluriprofessionnelle d'un centre commercial, sans être contraints par un seuil de population résidente. Des transferts d'officines pourront être autorisés vers un ensemble de communes contiguës listées par arrêté de l'ARS, dès lors que ces communes sont dépourvues d'officine, que l'une d'elles comprend au moins 2 000 habitants et que l'ensemble atteint le seuil de population global Ce choix d'un seuil de 2 000 habitants pour au moins l'une des communes a pour objectif d'assurer une offre pharmaceutique qui, d'une part, réponde aux besoins d'une population, et, d'autre part, garantisse les conditions de survie économique de l'officine sur ce territoire. D'ores et déjà, une première version de la méthodologie de zonage a été partagée et testée auprès de quatre ARS. La méthodologie nationale envisagée tient compte du rapport IGAS-IGF de 2016, confirmé par un rapport de la Cour des comptes, qui ont constaté un maillage officinal satisfaisant, avec 97 de la population vivant à moins de dix minutes en voiture d'une officine et 99,5 % à moins de quinze minutes. Ce constat partagé avec la profession nécessite de bien mesurer le choix de la maille, si vous me permettez l'expression, et des indicateurs consacrés. Le projet de décret relatif aux territoires fragiles vise ainsi à permettre aux ARS d'identifier, à partir de critères précis, les territoires pour lesquels l'accès à une pharmacie pour la population ne serait pas satisfaisant. L'évolution de la situation sanitaire devrait permettre de finaliser ces travaux réglementaires dans le courant de l'année 2022 avec l'ensemble des acteurs mobilisés. La parole est à M. Bernard Delcros,

compte aujourd'hui 25 pharmacies installées dans de petits bourgs ruraux et apportant une offre de services à un bassin de vie composé de 10 à 15 communes rurales autour de ce bourg-centre.

ces pharmacies seraient interdites d'installation. C'est bien la meilleure preuve qu'il faut revoir les conditions d'installation des pharmacies en milieu rural ! Je compte vraiment sur le Gouvernement pour tenir compte de cette réalité. Sachez que le maire et les élus de la commune de Vézac attendent

et de la santé. Madame la ministre, la fin du devait permettre de former plus de médecins. Mais la mise en oeuvre chaotique de la réforme des études de santé, l'insuffisance de places pour accueillir à la fois les redoublants de l'ancien système et les nouveaux entrants conduisent à une tout autre réalité. C'est en premier lieu insupportable pour les jeunes qui s'engagent dans des études de santé et voient leur parcours semé de tant d'embûches. Ils ont passé leurs examens dans le flou et l'incertitude, sans connaître le nombre de places ouvertes en deuxième année, sans savoir s'ils pourront continuer leur parcours ni où et comment. C'est en second lieu quand tant de nos territoires manquent de médecins et de professionnels de santé. L'université de Rouen voit ainsi le nombre de places en deuxième année de médecine augmenter de 6 % seulement- 9 % si l'on prend l'ensemble des filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie. On est loin des 14 % d'augmentation annoncés par le Gouvernement et encore plus de certaines universités parisiennes, alors que la Normandie est l'une des régions les plus déficitaires en médecins. Le Conseil d'État vient d'enjoindre à quinze universités, dont celles de Rouen et de Caen, d'augmenter de 20 % leurs capacités d'accueil. Pour ce faire, il leur faut impérativement des postes de chefs de clinique, par exemple, mais aussi de quoi réaliser des investissements.

ne comprenait aucun crédit supplémentaire en faveur des études de santé

qui grevait le nombre de professionnels de santé formés année après année. La question du nombre et de la répartition des professionnels de santé sur le territoire est donc une préoccupation majeure du Gouvernement. Pour l'année 2021,

Cette augmentation s'inscrit dans la trajectoire prospective proposée par la conférence nationale du 26 mars 2021 en remplacement du, au travers des objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former. Cette conférence, qui réunit l'ensemble des acteurs de la santé et les représentants d'élus locaux, a proposé de former 81 055 professionnels de santé, toutes filières médicales confondues, pour la période 2021-2025, soit une augmentation de plus de 14 % des effectifs sur cinq ans qui sera arrêtée par le Gouvernement. Pour la région Normandie, ce seront plus de 4 140

Leur planification pluriannuelle visera à mieux répondre aux besoins de santé identifiés à l'échelon de chaque région, tout en tenant compte des capacités de formation des universités et des centres hospitaliers universitaires. Cette augmentation ne se décrète pas simplement : nous devons accompagner la transformation des capacités d'accueil et de formation hospitalière pour donner corps à notre ambition. Cela ne peut se faire, vous en conviendrez, qu'en maintenant la qualité de ces formations, qui nécessitent un haut niveau d'exigence. Par ailleurs, en plus du pilotage territorial, nous maintiendrons des objectifs nationaux pour disposer d'une capacité de suivi quantitatif. quantitatif. Notre action en matière de régulation s'apprécie également à travers l'ouverture des postes d'internat. Depuis 2017, nous opérons un rééquilibrage territorial en augmentant chaque année le nombre de postes offerts dans les régions les moins bien dotées en médecins, tout en stabilisant les effectifs dans les régions les mieux dotées.

En zone rurale, faire constater un décès par un médecin devient un exercice de plus en plus difficile, en particulier le week-end et les jours fériés, où le manque de médecins disponibles est encore plus flagrant. Le 15 avril dernier, le maire de la commune de Les Salles, dans mon département, M. Jean-Hervé Peurière, a vécu cette expérience très difficile et désagréable. Entouré de pompiers et de gendarmes, après avoir contacté, pendant plusieurs heures, cinq cabinets médicaux, le médecin du SMUR (structure sans aucun résultat, il a dû appeler son médecin personnel pour faire constater le décès d'une personne de 81 ans. Face à cette situation, les maires sont en première ligne et sont régulièrement interpellés par leurs administrés. Ils se retrouvent seuls, souvent démunis, confrontés à des situations humaines extrêmement douloureuses et compliquées à gérer. La seule solution possible est actuellement de procéder à une réquisition administrative, procédure exceptionnelle et lourde pour un élu local. Cette responsabilité pesante pour les maires n'est satisfaisante ni humainement ni juridiquement. De plus en plus d'élus souhaitent l'évolution des modalités de constatation d'un décès en cas d'absence d'un médecin disponible sur un territoire, et ce dans des délais raisonnables. Certains proposent de faire exceptionnellement appel aux pompiers ou aux infirmiers. Ce serait aussi une avancée considérable pour les familles, qui, dans ce moment de deuil, ne comprennent pas ces carences. Ainsi, madame la ministre, je souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter pour répondre aux préoccupations des élus et à la souffrance des familles. La parole est à Mme la ministre

de décès- médecins retraités, étudiants de troisième cycle ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent, praticiens à diplôme étranger hors Union européenne, à compter de la deuxième année de leur parcours de consolidation. Cette extension permet de répondre à un double enjeu : celui d'une diversification des personnes susceptibles d'être présentes sur le territoire tout en respectant le caractère médical d'un certificat de décès. L'établissement de L'établissement de ce certificat suppose en effet un diagnostic sur les causes de décès après examen du corps du défunt. Ce diagnostic est d'autant plus important qu'il est utilisé pour la veille sanitaire. Les données figurant sur les certificats de décès sont utilisées pour établir les statistiques de décès et servent à identifier des alertes de santé publique de nature à appeler des mesures de la part des autorités sanitaires nationales ou régionales. Il emporte également des conséquences sur les opérations funéraires dans la mesure où un obstacle médico-légal peut venir les retarder. Les médecins sont formés à évaluer la présence ou non d'un obstacle médico-légal, ce qui n'est pas le cas des pompiers ou des infirmiers. Pour l'ensemble de ces raisons, une évolution nouvelle des catégories de professionnels susceptibles d'établir un certificat de décès n'est pas actuellement envisagée. Cependant, le ministère des solidarités et de la santé est à l'écoute de toutes les propositions constructives

Cette décision reposait sur une hypothèse sanitaire, qui n'a pas donné lieu à réévaluation. Depuis, de nombreuses études sont parues sur le sujet. Les enfants d'âge primaire participent très faiblement à la circulation du virus. Les clusters sont surtout familiaux et non scolaires, comme l'ont confirmé les campagnes de tests. Sans compter les difficultés de port du masque à cet âge. A-t-on pris en compte ces éléments ? Les professionnels de l'enfance alertent et s'interrogent. Une étude allemande du 30 juin dernier a mis en évidence des taux de CO2 expiré après port du masque de cinq à six fois supérieurs à la normale. Quel impact sur le cerveau en construction de nos enfants ? Pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, ORL, ophtalmologistes relatent divers troubles de la croissance et pathologies dus au port quotidien du masque par un enfant en développement. Enfin, le masque met en difficulté les élèves les plus fragiles, inhibe les interactions entre enfants et est pourvoyeur de retards d'apprentissage pour la lecture et l'écriture. Voix forcée, baisse de l'écoute et de l'intelligibilité, altération de la conscience phonologique, somnolence sont le quotidien de nos enfants. Tout cela a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact pluridisciplinaire ? Compte tenu des enjeux de développement de toute une génération, les sociétés savantes de pédiatrie ont appelé, le 17 juin dernier, à une fin d'année à visage découvert sans être entendues, alors même que nos voisins belges et anglais, à circulation virale plus intense, ont statué- avec réactivité -sur la suppression du masque pour les enfants à l'école primaire dès le printemps. Ne pourrait-on imaginer une politique de bon sens, qui ajuste le port du masque en fonction de la saisonnalité du virus ? En outre, en cas de pic épidémique, des campagnes de dépistage salivaire territorialisées permettraient de limiter le masque aux seules classes touchées. La covid et tous ses variants ne sont pas des maladies pédiatriques. Les adultes doivent protéger les enfants et non faire peser sur ces derniers le soin de leur protection, et ce d'autant moins que nous disposons maintenant de différents moyens de lutter contre le virus. Madame la ministre, quelle sera la politique du Gouvernement en matière de port du masque à l'école primaire pour la rentrée prochaine ? J'espère votre réponse courageuse ; elle est attendue par des millions de Français. Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Kristina Pluchet, depuis septembre 2020, les élèves ont été accueillis au sein des écoles maternelles et élémentaires dans le respect du protocole sanitaire élaboré sur la base des avis du Haut Conseil de la santé publique. Depuis le début de la crise sanitaire, notre ligne de conduite vise non seulement à protéger, mais aussi à permettre le plus possible la scolarisation des élèves, en particulier des plus jeunes. Pour tâcher de concilier ces impératifs, une foire aux questions a été établie pour adapter la mise en oeuvre du protocole sanitaire dans chaque territoire, en fonction de la configuration des établissements et de la situation sanitaire locale. Ce choix de garder les classes ouvertes, dans la mesure du possible, selon l'intensité de circulation du virus, et la mobilisation de tous les acteurs ont permis à l'ensemble des élèves du primaire de bénéficier des enseignements en présentiel. La continuité a permis d'atténuer l'impact des confinements et restrictions depuis le début de la crise. Le ministre de l'éducation nationale nous confirme que les résultats des évaluations nationales mi-CP et CE1 témoignent de l'effet positif de cette décision. Face à la circulation du virus et à l'apparition de différents variants plus contagieux, tous les moyens ont été mobilisés : réalisation de tests salivaires, respect des distanciations sociales, port du masque en classe. Le risque avéré de transmission du virus entre les enfants demeure, particulièrement dans les écoles, qui sont des lieux clos des zones de brassage de la population. Tant la Société française de pédiatrie, en accord avec les recommandations de l'OMS, que le Haut Conseil de la santé publique se sont prononcés en faveur du port du masque pour les enfants de plus de 6 ans. Dans son avis du 29 octobre 2020, le Haut Conseil a souligné qu'il n'existe pas de contre-indications dermatologiques, pneumologiques, ORL, phoniatriques ou psychiatriques au port du masque. Pour autant, l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires n'est pas absolue. Les élèves de l'école maternelle, en plein apprentissage du langage, n'en portent pas, et des masques inclusifs ont été mis à disposition de leurs enseignants. Un décret prévoit également des exceptions sur avis médical, notamment pour les enfants en situation de handicap. Par ailleurs, lors de la prise des repas, de la pratique d'une activité sportive, le port du masque n'est pas obligatoire. Dans ces situations, une attention particulière est portée à la limitation du brassage. À ce jour, le développement rapide du variant delta ne nous permet pas d'apprécier précisément la situation de la rentrée scolaire prochaine. Le protocole sanitaire au sein des écoles sera adapté en fonction de la situation que nous connaîtrons. Plusieurs scénarios pédagogiques sont d'ores et déjà élaborés afin d'organiser la rentrée des élèves de la façon la plus sereine possible. De nouveau, notre priorité est double, et je pense que vous en partagerez les objectifs : allier sécurité sanitaire et ouverture des écoles. Jusqu'ici, le pari est tenu, notre pays ayant maintenu ses classes plus ouvertes que nombre de nos voisins.

Il comportait une classification des pays en trois catégories, selon qu'ils recevaient ou non le vaccin. Qu'en est-il de cette liste ? Le ministère des affaires étrangères ne nous l'a toujours pas transmise.

Les ministres Le Drian et Lemoyne, qui m'ont demandé de vous répondre, sont particulièrement investis sur le déploiement de notre stratégie vaccinale. Je voudrais rappeler tous les efforts que la France déploie depuis le début de la crise pour que la vaccination soit accessible à tous et dans tous les pays- en somme, pour faire de ce vaccin un bien public mondial. La solidarité vaccinale, dont la facilité Covax est la meilleure incarnation, est un impératif moral, mais aussi la seule façon de mettre fin, ensemble, à la pandémie. c'est un principe intangible, la France est aux côtés de ses citoyens, où qu'ils soient dans le monde. Elle est le seul pays à avoir lancé la vaccination de ses communautés à l'étranger, là où n'existe pas de solution locale de vaccination avec des vaccins reconnus par l'Agence européenne des médicaments. En comparaison, certains de nos partenaires européens et internationaux ont des plans de vaccination, certes, mais uniquement pour leurs agents publics expatriés. Dès le mois de décembre dernier, nous avons lancé des travaux en ce sens, avant même que la vaccination ne démarre sur le territoire national.

Jusqu'ici, cette vaccination a été organisée en s'appuyant sur les ressources propres des ambassades et des consulats généraux, avec l'appui de structures sanitaires locales partenaires. Comme vous le savez, il s'agit d'opérations logistiquement lourdes et complexes, qui supposent l'accord des pays dans lesquels elles sont réalisées. Les autorisations ne sont parfois pas encore données et nous travaillons activement avec ces pays pour résoudre les freins dans les meilleurs délais. Par ailleurs, conjointement avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, nous allons amplifier nos efforts dans les semaines à venir, en lien avec l'élargissement de la politique vaccinale nationale. L'avis de la Haute Autorité de santé du 9 juillet dernier sur la vaccination des Français de l'étranger avec le vaccin Janssen nous invite à nous inscrire à la fois dans une géographie plus vaste et dans une autre temporalité. En outre, lors de leur passage en France, par exemple pour leurs congés, cet été, nos compatriotes de l'étranger peuvent tous se faire vacciner gratuitement. Je rappelle que les délais d'injection entre deux doses ont été réduits plus court, à savoir 21 jours, ce qui permet un recours le plus vaste possible à cette opportunité pour nos concitoyens résidant le reste de l'année à l'étranger. Ceux de nos compatriotes qui reviennent d'un pays en liste rouge et qui seraient soumis à une quarantaine administrative, et non à un isolement,

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaitais vous alerter sur les difficultés rencontrées par les élus locaux dans l'interprétation et l'application de leur avis d'arrêt de travail pour congé maladie. De nombreux élus, de bonne foi, convaincus de pouvoir continuer à exercer leur mandat, se voient réclamer le remboursement intégral des indemnités perçues au titre de leur travail salarié pour seulement quelques heures passées à exercer un mandat local- et, comme vous le savez, pour une indemnité de quelques euros seulement ... En effet, très peu d'élus savent qu'ils doivent préalablement solliciter auprès de leur médecin une autorisation spécifique d'exercer une fonction élective pendant le congé maladie. Il est d'ailleurs important de noter que les praticiens eux-mêmes ne sont bien souvent pas au courant de cette subtilité, contrairement à ce que prétend la Caisse nationale de l'assurance maladie Il n'est pas acceptable que ces élus, qui ne comptent pas leurs heures au service de leurs concitoyens, soient sanctionnés de la sorte, d'autant que les voies de recours sont limitées.

L'année dernière, le Gouvernement avait reconnu un défaut d'information des élus et des médecins. La CNAM avait annoncé une campagne de communication à destination des praticiens, ainsi qu'une évolution de la rédaction du formulaire Cerfa d'avis d'arrêt de travail, avec l'apparition distincte d'une mention autorisant l'activité de l'élu local, à l'instar des dispositions existantes en matière d'horaires de sortie. Malheureusement, force est de constater que la situation n'a pas changé. Les exemples récents d'élus qui se heurtent à l'inflexibilité de l'administration sont encore trop nombreux. Il paraît donc urgent de concrétiser les engagements pris.

du code de la sécurité sociale : le salarié placé en congé maladie doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, un salarié par ailleurs élu local placé en congé maladie ne peut régulièrement exercer son mandat électif que si son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Dans le cas contraire, il peut se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, la Cour de cassation assimilant les indemnités de fonction à une rémunération d'activité. Cette difficulté, que des élus de toute bonne foi ont pu rencontrer, a été soulignée par les travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Elle était le fruit d'un défaut d'information des élus sur la nécessité de préciser à leur médecin de mentionner, le cas échéant, qu'ils sont autorisés à exercer leur mandat électif pendant leur arrêt de travail. Cette réglementation a déjà fait l'objet d'un

si un patient ne prévient pas son médecin qu'il est également élu local, le médecin n'indiquera pas, de toute bonne foi lui aussi, l'incompatibilité de l'état de son patient avec son mandat, ou les réserves partielles qu'il pourrait y opposer. C'est alors la responsabilité du médecin qui serait engagée. Pour répondre de façon efficace à ce problème, nous avons cherché à mieux informer les élus sur leurs droits

Si chacun peut comprendre qu'il faut éviter la fraude et produire des certificats de vie ou attestations d'existence, les tracasseries administratives et refus de certificats de vie pourtant valables entraînent des suspensions indues de versement de retraite. Pourtant, nos compatriotes établis à l'étranger soulignent souvent qu'ils envoient leurs certificats de vie ou attestations d'existence par la poste et par voie électronique, parfois à plusieurs reprises. Malgré cela, des difficultés demeurent et ils ne touchent pas un centime de leur retraite. La mise en place récente d'un centre unique pour toutes les réclamations devrait apporter quelques améliorations, mais de grands problèmes demeurent. En ce qui concerne les futurs retraités, on constate également de nombreux cas de blocages ou de retards importants dans le traitement des rachats de trimestres des périodes à l'étranger.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) se doit de leur proposer un devis correspondant aux trimestres rachetables. Or les demandes restent sans réponse- dans certains cas, depuis des mois. Monsieur le secrétaire d'État, pour traiter ces multiples retards, ne peut-on envisager un renforcement de personnels au groupement d'intérêt public Union Retraite

secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Ronan Le Gleut, vous interrogez le Gouvernement sur le délai de traitement par la CNAV des dossiers de Français établis hors de France pour la liquidation des retraites,

observé une hausse des demandes de plus de 50 % au premier semestre 2021 par rapport à l'année précédente. Des plans d'action sont actuellement déployés pour le traitement de ces demandes. L'ensemble des leviers à disposition de la CNAV sont mobilisés formation d'agents redéployés, recours à des CDD, augmentation du nombre d'heures supplémentaires, voire modification des méthodes de traitement. Plus globalement, le Gouvernement, bien conscient du problème, a saisi la CNAV depuis plusieurs mois pour améliorer sa qualité de service. Nous souhaitons en effet réduire les délais de traitement, mais aussi assurer la justesse du calcul de la pension, qui est parfois particulièrement complexe,

Nous avons des témoignages de femmes et d'hommes qui ne touchent plus un centime de retraite. Puisque vous reconnaissez ces retards, il faut agir vite et fort ! La parole

Il est aujourd'hui un bien triste constat : notre langue française est étrillée par l'écriture dite inclusive. En effet, un nombre croissant d'établissements universitaires contreviennent à la circulaire du 21 novembre 2017, en usant du point médian ou de la syntaxe dite épicène. Parmi eux - la liste n'est pas exhaustive -, la faculté de droit de Nanterre, où les panneaux d'affichage, les mails de la présidence ou des supports de travaux dirigés Paris Dauphine, où ce sont les sujets de partiels ou les polycopiés de cours qui sont touchés. Ce phénomène concerne à la fois des communications internes adressées aux étudiants et des publications destinées au public. Mais il y a plus grave encore : des rapports publiés par un certain nombre d'institutions relaient eux aussi cette orthographe néfaste. en février 2019, le Conseil d'État avait rejeté un recours soumis à son appréciation et confirmé l'esprit de la circulaire Philippe, en enjoignant aux administrations de respecter les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur dans la rédaction de leurs actes administratifs. Cette jurisprudence ne doit pas être minimisée, car elle vient consacrer les conclusions d'un rapport de l'Académie française mettant en garde depuis près de trois ans contre « un péril mortel pour la langue nationale de l'éducation nationale, a étendu l'interdiction de l'écriture inclusive aux usages pédagogiques. C'est une avancée louable, mais encore insuffisante, alors qu'un nombre substantiel d'administrations, de rectorats ou de directions d'établissements publics d'enseignement s'en exonère. Vous inaugurerez en mars prochain la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, où fut prise l'ordonnance généralisant l'utilisation du français dans les actes administratifs. c'est précisément par ces actes administratifs que l'écriture inclusive bafoue aujourd'hui notre héritage culturel. Au regard de la violation flagrante de la circulaire Philippe, n'est-il pas temps d'initier une réponse législative pour consacrer définitivement les principes posés par notre académie ? C'est un patrimoine sensible que nous avons à préserver. Comme l'écrivait la philosophe Simone Weil, « nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. » Il en va de même pour notre langue, aujourd'hui en péril.

Avec la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 que vous avez citée, le Gouvernement a clairement rappelé les principes de rédaction des textes officiels. Cette circulaire invite au maintien des règles en usage, qu'elles soient typographiques, par l'exclusion du recours aux formes abrégées par un point médian ou par tout autre séparateur graphique faisant ressortir l'existence d'une forme féminine en complément de la forme masculine, ou grammaticales, avec le masculin comme forme neutre. Les administrations de l'État doivent se conformer à ces règles, pour des raisons d'intelligibilité et de clarté, non seulement parce que la complexité de la typographie dite inclusive pénalise les personnes affectées d'un handicap, mais aussi parce que la majorité de nos concitoyens en ignore les mécanismes et ne reconnaît plus d'ailleurs sa propre langue. L'apprentissage et la maîtrise de la langue française relevant des missions fondamentales de l'école, il était important que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rappelle les principes de rédaction dans la circulaire du 5 mai 2021, adressée aux rectrices et aux recteurs d'académie, aux directrices et directeurs de l'administration centrale et à leur personnel. La langue française apprise et pratiquée par les élèves et les lycéens reste soumise à la règle commune. L'exclusion de la typographie inclusive ne saurait cependant accréditer l'idée que la langue française conforte les inégalités entre les femmes et les hommes. Nous devons renforcer notre engagement pour l'égalité, et privilégier les recommandations de la circulaire du 21 novembre 2017 en faveur de la féminisation de notre langue. Cela passe notamment par la promotion du recours à la féminisation systématique des noms de métier ou de fonction exercés par une femme ou à des mots épicènes. L'application systématique de ces préconisations, qui accorde aux femmes, à l'écrit comme à l'oral, autant de visibilité et d'égards qu'aux hommes, contribue à la consolidation et à l'évolution de la langue française, sans pour autant la dénaturer.

Cependant, le virus menace toujours, notamment depuis l'apparition du variant Delta, plus contagieux, en particulier dans les lieux clos. Le constat est simple : malgré l'accélération de la vaccination, il nous faudra désormais apprendre à vivre avec la covid et ses variants pour les années à venir. Pour faciliter l'organisation du secteur culturel et de l'événementiel, des solutions innovantes émergent. Parmi elles, je veux citer l'expérimentation menée par le centre de congrès et d'exposition de Labège, Diagora, en Haute-Garonne, dans mon département, en partenariat avec Dassault Systèmes, sur l'analyse des flux d'air et la simulation numérique pour la réouverture des salles de spectacles et d'événementiel. Ce dispositif, développé par un jeune ingénieur toulousain, s'appuie sur le logiciel de Dassault Systèmes, déjà utilisé par plusieurs hôpitaux à travers le monde Cette expérimentation permettrait que les lieux culturels puissent accueillir du public dans les meilleures conditions, avec des mesures sanitaires adaptées et des conditions de placement scientifiquement démontrées. Cette solution innovante permettrait non seulement d'améliorer la sécurité des spectateurs avec une ventilation optimisée, mais également de répondre à la souffrance du secteur culturel sur l'ensemble de notre territoire. Elle consiste à construire un « jumeau numérique » de la salle pour y étudier les flux d'air. Ces derniers sont ensuite modifiés en fonction des résultats, afin d'empêcher qu'ils atteignent les personnes dans la salle. Il ne serait ainsi plus nécessaire d'instaurer une jauge limitant le nombre de spectateurs présents. Ce dispositif serait une mesure complémentaire au passe sanitaire actuellement en vigueur et garantirait une assurance supplémentaire pour les spectateurs. Pour que cette expérimentation puisse aboutir, il est nécessaire de l'élargir au plus grand nombre d'acteurs culturels et événementiels, afin de leur permettre de reprendre au plus vite leurs activités de manière pérenne.

secrétaire d'État. Madame la sénatrice, le Gouvernement a été particulièrement mobilisé sur cet enjeu des expérimentations dans les salles de spectacles et de concerts dès le début de l'année 2021.

au sein des salles de spectacles et ainsi à contribuer à la définition de protocoles sanitaires transposables à grande échelle. De nombreuses collectivités se sont manifestées pour organiser ces expérimentations. Vous avez cité l'exemple de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, Sicoval, dans votre département de la Haute-Garonne. Je le souligne, elles demandent demandent des mois de préparation, un soutien financier conséquent et, surtout, des protocoles scientifiques particulièrement complexes. À ce jour, une seule a pu avoir lieu à l'occasion du concert d'Étienne de Crécy et du groupe Indochine, le 29 mai dernier à l'Accor Arena de Paris. publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le dispositif sanitaire a permis à 5 000 personnes d'y assister. Les résultats de l'étude rendus publics la semaine dernière par l'AP-HP sont très encourageants, puisque les scientifiques considèrent qu'il n'y a pas eu de surrisque pas eu de surrisque de transmission du covid-19 pendant le concert. Ces résultats doivent pouvoir être également analysés par le ministère de la santé et l'ensemble des autorités sanitaires. Ces expérimentations étaient, je crois, utiles dans cette période d'attente de la reprise. Vous le savez, les salles de spectacles et de concerts ont ont pu rouvrir leurs portes le 19 mai dernier et les restrictions de jauges ont été levées depuis le 1juillet. Nous avons mis en place des règles sanitaires strictes, pour que cela se passe dans les meilleures conditions possible, notamment avec la mise en place du passe sanitaire,

Le ministère de la culture reste évidemment en dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. L'enjeu est de mieux comprendre et de mieux maitriser tout ce qui peut avoir une influence sur la transmission du virus, notamment les flux d'air dans les lieux culturels. La parole est à Mme Émilienne Poumirol,

M. le ministre de l'intérieur. Madame la ministre, en novembre dernier, après une longue gestation, le Livre blanc de la sécurité intérieure était enfin dévoilé. Une proposition figurant dans le titre intitulé « Renouveler le pacte de protection et de sécurité » a retenu toute mon attention, et suscite surtout beaucoup d'inquiétude. Il est proposé de définir une nouvelle méthode pour partager sur le territoire national les compétences de la police et de la gendarmerie. Pour mémoire, selon la règle en vigueur, la responsabilité de la police nationale dans une commune est soumise au cumul de deux critères : une population supérieure à 20 000 habitants et une délinquance ayant les caractéristiques de celle des zones urbaines. Le Livre blanc préconise une évolution de ce seuil de population. Au-dessous de 30 000 habitants, le principe serait de confier le territoire à la gendarmerie.

Mécaniquement, les départements les plus ruraux se verraient donc totalement exclus des zones de la police nationale, y compris pour leur chef-lieu. La Haute-Saône serait placée dans un tel cas, ce qui ne manque pas de raviver l'inquiétude des personnels du commissariat de Vesoul, qui sont exposés depuis plusieurs années à des incertitudes récurrentes. Je ne doute pas de l'opportunité de faire évoluer les critères de répartition des forces de sécurité et je partage l'ambition de passer d'un « modèle quantitatif » à un « modèle qualitatif reposant sur une analyse locale, pragmatique et objective

Je vous remercie d'avance, madame la ministre, de m'expliquer cette contradiction et, surtout, les critères objectifs sur lesquels se fonderait cette réorganisation, qui ne doit avoir qu'un seul but : assurer à tout citoyen un service de sécurité publique le mieux adapté aux réalités du territoire sur lequel il se trouve.

déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Olivier Rietmann, apporter des réponses concrètes aux problèmes de délinquance et d'insécurité de nos concitoyens exige des moyens. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat

pour une adaptation constante aux évolutions de la délinquance, pour répondre à l'objectif majeur du renforcement de la présence sur la voie publique et pour donner aux policiers et gendarmes les moyens d'assumer leurs missions dans les meilleures conditions d'efficacité possible. La police nationale a d'ores et déjà accompli ou engagé d'importantes réformes en la matière. Je pense ainsi à la création d'échelons zonaux en sécurité publique et en police judiciaire et à l'expérimentation, dans trois départements, de directions départementales de la police nationale. Les coopérations et complémentarités entre la police et la gendarmerie, notamment la répartition de leurs forces sur le territoire, constituent également un enjeu important de notre dispositif de sécurité et un sujet auquel sont particulièrement attentifs les élus locaux.

entre la police et la gendarmerie entre 2002 et 2014 pour adapter leur organisation aux évolutions de l'urbanisation et de la délinquance, accroître l'homogénéité des zones de compétence et permettre aux deux forces de renforcer leur complémentarité et d'optimiser

et de gendarmerie. Cette ouverture fait écho au Livre blanc de la sécurité intérieure, qui préconise de mieux faire coïncider la répartition des forces avec les caractéristiques spécifiques de chaque territoire. M. le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à la direction générale de la police nationale

pour être pleinement efficace, de la transparence et de la pédagogie. Or, bien que nous puissions pleinement partager l'objectif de limiter les risques pour les usagers de la route, les mesures que vous avez prises concernant la généralisation à l'ensemble du territoire national des voitures radars banalisées par des opérateurs privés manque de transparence. Où est la transparence, face à l'absence de toute communication sur les résultats obtenus en termes d'amélioration de la sécurité routière ? Où est la transparence, face à l'absence d'un calendrier clair et d'une méthode explicitée ? est la transparence, face à l'absence de garanties sur les contrôles de ces opérateurs ? Je pense aux témoignages inquiétants d'automobilistes sur des dérives constatées par certaines compagnies visant à les piéger pour les inciter à franchir les limitations de vitesse,

Sans transparence et sans pédagogie, les Français voient cette nouvelle mesure comme un nouvel impôt déguisé, un moyen pour l'État de remplir les caisses sur leur dos, d'autant que, si l'on en croit différentes projections, on passerait de 1,5 million de PV à 12 millions. Ils y voient le symbole d'une politique de sécurité routière ayant définitivement basculé dans le tout répressif. Ils y voient enfin, et surtout, une nouvelle rupture d'égalité entre les urbains et ceux qui habitent dans les territoires ruraux, ces derniers n'ayant d'autres choix, pour se déplacer, que d'utiliser leur voiture chaque jour. Abaissement Abaissement de la vitesse sur les routes secondaires à 80 kilomètres par heure, puis rétropédalage, augmentation des radars tourelles, qui ne sont pas toujours signalés dans mon département, et, enfin, voitures radars banalisées par des opérateurs privés. Cela commence à faire beaucoup, y compris pour les plus conciliants ! Prenez garde, madame la ministre, à ne pas souffler sur les braises. madame la ministre,

Les premières voitures radars banalisées ont progressivement été déployées à compter de 2013. Avant le lancement, en 2018, de la mesure d'externalisation, on en comptabilisait 383, exclusivement conduites par des policiers ou des gendarmes. Depuis 2018, le déploiement progressif de voitures radars à conduite externalisée, au nombre de 145 à ce jour, a entraîné la suppression de 116 voitures radars, qui seront, à terme, toutes remplacées.

le chiffre de 12 millions de PV n'est fondée sur aucun constat. Aujourd'hui, la mesure d'externalisation de la conduite des voitures radars permet d'accroître l'utilisation des voitures, sans pour autant engendrer une multiplication des PV. S'agissant de la pertinence de mettre en place un système d'identification des voitures radars à conduite externalisée,

: des actes malveillants à leur égard sont régulièrement constatés dans les régions concernées, prenant parfois la forme d'actes dangereux, dont certains ont donné lieu à dépôt de plainte ou de main courante. M. le ministre de l'intérieur a demandé à ses services d'étudier la pertinence d'une publication par les préfectures, sur leur site internet, de la cartographie des axes contrôlés par ces véhicules, comme l'ont déjà fait les préfectures de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Enfin, monsieur le sénateur, vous affirmez que l'État utilise ces dispositifs pour alimenter son budget, sans gain pour la sécurité routière. C'est une inexactitude démentie par les documents par les documents budgétaires transmis chaque année au Parlement : on y découvre, d'une part, que l'argent des radars est utilisé à plus de 85 % en faveur de la sécurité routière dans le cadre d'un compte d'affectation spéciale

En effet, cette fusillade a entraîné l'intervention du seul et unique équipage de nuit du commissariat de Gap. Oui, madame la ministre, la sécurité nocturne de Gap, préfecture des Hautes-Alpes, et de ses 42 000 habitants, repose sur un équipage. Il ne s'agit malheureusement que de la partie émergée de l'iceberg de la sécurité. En effet, la réduction structurelle des effectifs a pour conséquence une dégradation des conditions de travail des personnels de police et un service rendu à la population d'une qualité moindre. Alors que le commissariat de Gap comptait 64 personnes en décembre 2018, ils ne sont plus que 51 en 2021. Ce sous-effectif de fonctionnaires de police rend impossible la mission de sécurité que l'on doit aux Gapençaises dans le même temps, la délinquance ne cesse de croître à Gap, et les manifestations sur la voie publique y ont été multipliées par cinq en moins de trois ans. La conséquence directe de cette situation tendue est une baisse de l'attractivité des postes, la moyenne d'âge des policiers de Gap étant de 48 ans, soit deux fois moins, en région parisienne. Outre les problèmes d'effectifs, les locaux du commissariat de Gap manquent d'entretien et sont vétustes. À titre d'exemple, sachez, madame la ministre, que les vestiaires des agents féminins ont été installés dans des locaux précédemment occupés par les véhicules de service Comment peut-on traiter nos forces de l'ordre de cette manière, pour ensuite leur demander de risquer leur vie au quotidien pour protéger nos populations ? Certes, les Hautes-Alpes ne représentent que 0,20 % de la délinquance nationale. Pour autant, nos concitoyens méritent d'être traités de la même manière que dans les grandes agglomérations.

Que comptez-vous faire, madame la ministre, face au manque de fonctionnaires de police à Gap ? Allez-vous enfin renforcer les effectifs comme il est demandé ? Quels seront précisément les moyens alloués à ce commissariat en termes d'investissements ? La parole est à Mme la ministre

L'arsenal législatif se renforce et s'adapte, avec la récente proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais aussi avec les lois portées par mon collègue garde des sceaux. Le Beauvau de la sécurité

de faire reculer la délinquance. J'en viens maintenant au coeur de votre question, monsieur le sénateur, qui concerne la ville de Gap. La sécurité publique, notre police de la sécurité du quotidien, y dispose d'un effectif opérationnel qui a augmenté de 10 depuis le début du quinquennat, pour atteindre à ce jour 53 gardiens de la paix. Je tiens à préciser, monsieur le sénateur, que Gap se trouve ainsi en situation favorable par rapport à d'autres circonscriptions de sécurité publique comparables.

devrait conduire, à terme, à des modifications dans l'occupation de la cité administrative. La sécurité publique devrait à cette occasion gagner de l'espace supplémentaire, par exemple pour accueillir le service départemental du renseignement territorial. Monsieur le sénateur, qu'il s'agisse des conditions de travail des policiers ou des moyens qui leur sont nécessaires pour accomplir efficacement leurs

Les fortes précipitations et les orages intervenus voilà quelques semaines dans le Val-de-Marne ont provoqué des inondations sur la RN 19, entre Boissy-Saint-Léger et Bonneuil-sur-Marne, dans le tunnel. L'axe a été rapidement infranchissable, piégeant plusieurs automobilistes et saturant la circulation sur cette zone. Hélas, ce n'est pas une première, puisque deux inondations quasiment similaires étaient survenues en 2020, avant que ne soit ouverte, en avril 2021, la déviation de La RN 19 est une artère très empruntée par les Franciliens. Or il semble que, aujourd'hui, pluie rime inéluctablement avec inondation. Certes, la forme de cuvette de cette section n'aide naturellement pas l'eau à s'évacuer, mais les défaillances répétées du système de pompage sont aussi en cause. Sur place, les élus évoquent une erreur de conception et l'absence d'une retenue d'eau capable de faire face aux forts orages. Si la direction des routes de l'Île-de-France semble résignée face à ces situations, tel n'est pas le cas des élus.

de la station. Concrètement, il s'agit de mettre définitivement hors d'atteinte des équipements électriques qui se montreraient vulnérables par forte pluie. Afin d'assurer la pérennité des dispositifs mis en place, la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France va accroître ses efforts de maintenance et de surveillance de la station de pompage. L'État est pleinement conscient

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la question de la prise en compte des cellules pénitentiaires dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). cette loi de décembre 2000 prévoit l'obligation pour certaines communes de disposer d'un nombre minimal de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel.

à inclure les cellules d'établissements pénitentiaires dans le décompte des logements sociaux des communes. L'implantation d'une prison est en effet une décision unilatérale de l'État et n'est pas sans conséquence sur la vie de la commune ; les impacts

puisque les détenus sont comptabilisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la population légale de la commune. Cette comptabilisation peut avoir pour conséquence de faire franchir des seuils démographiques impliquant de nouvelles obligations.

L'État intègre déjà dans l'inventaire des logements locatifs sociaux un certain nombre de structures collectives d'hébergement spécialisé telles que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les logements pour étudiants saisonniers, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'accueil de demandeurs d'asile.

tous les ménages sous plafond de ressources. Il est donc en tout état de cause évident que la finalité des établissements pénitentiaires ne saurait être assimilée à celle du logement social. Je rappelle que le parc social loge aujourd'hui un Français sur six et que, deux millions de demandeurs de logements sociaux étant en attente, les besoins restent importants. Le Gouvernement a

subissait l'effondrement d'un tunnel sur l'un de ses ruisseaux dits couverts. Cet effondrement a engendré un cratère de quarante mètres de diamètre, emportant une aire de jeux pour enfants, un terrain de tennis et une partie du terrain de football Ces tunnels, qui sont présents dans bien d'autres communes gardoises, avaient été édifiés sur des ruisseaux afin de créer des plateformes suffisamment vastes pour y accueillir des infrastructures inhérentes à l'activité minière. Malheureusement, lorsque les exploitants ont mis fin à leur activité, ils ont suivi une procédure prévue par une réglementation qui ne prenait pas en compte ces ouvrages. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que ces tunnels sont de véritables menaces pour les habitants vivant à proximité, ni que ces ouvrages étaient bel et bien inhérents à l'activité minière. À la fermeture des mines, nationalisées depuis 1946, l'État a vendu une grande partie de ses terrains. Ainsi les acquéreurs, qu'ils soient publics ou privés, ont-ils hérité, sans être en mesure d'en être parfaitement conscients, des contraintes afférentes au droit du sol. les particuliers ni les communes ne peuvent assumer seuls la prise en charge des dépenses liées à la sécurisation de ces ouvrages gigantesques. Depuis l'effondrement évoqué,

pas fait l'objet d'un encadrement réglementaire au titre du code minier. Ces ouvrages relèvent bien de la responsabilité des personnes qui ont souhaité en récupérer la propriété. Ainsi les droits et responsabilités afférents, notamment les travaux de réhabilitation et d'entretien que vous évoquez, reviennent-ils aux actuels propriétaires, souvent des communes, dont les moyens techniques et financiers sont parfois limités. tenu des faibles ressources financières de ces propriétaires, des modalités d'accompagnement au titre de la solidarité nationale sont mises à l'étude- une participation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fameux fonds Barnier,

souhaite vous interroger sur la façon dont le Gouvernement compte intervenir au soutien des acteurs ayant fait le choix de développer un hydrogène vert, notamment dans les territoires.

Dans ce secteur, la France a clairement choisi de développer la filière électrolyse, un objectif ambitieux de 40 gigawatts en 2030 étant défini. Les territoires, acteurs incontournables d'un maillage efficient, ont pareillement pris le sujet

Plus performant qu'un électrolyseur et plus rentable qu'une éolienne, le procédé de gazéification à très haute température est duplicable et adaptable partout dans les territoires ruraux. Par ailleurs, cette pratique, qui n'entre pas en concurrence avec les cultures vivrières, nettoie les sols, purifie les nappes phréatiques, capte massivement du CO2 par photosynthèse et augmente de 10 à 15 % le rendement des cultures suivantes. Cette technique est un véritable challenge qui nécessite avant tout alliances et synergies entre autorités publiques nationales et locales, entreprises, organisations de la société civile et autres parties prenantes. Aussi, à l'heure où les différents plans sectoriels de relance gouvernementaux se multiplient, quelle est la place réservée à cette technique importante dans le déploiement stratégique du plan hydrogène vert en France ?

de composants clés, sur la mobilité lourde ou sur la décarbonation de l'industrie. Tout cela représente un montant de 1,5 milliard d'euros d'aides pour la France. Le projet que vous évoquez plus particulièrement, porté par Quairos Énergies, vise à l'installation d'une usine de gazéification de chanvre sur le territoire de Trangé dans le cadre de l'appel à projets « Briques technologiques

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les inquiétudes soulevées par la multiplication des projets d'implantation de parcs éoliens dans les territoires ruraux, en particulier dans le Cantal. S'inscrire dans une logique de croissance des énergies renouvelables, j'y suis favorable, bien évidemment. En revanche, le faire de manière durable, harmonieuse et réfléchie serait un gage de confiance adressé aux élus de nos territoires, à nos concitoyens et à l'ensemble des acteurs économiques et agricoles. Il est toujours paradoxal de voir débarquer à la hussarde des entreprises démarchant nos territoires, exigeant des rémunérations mirobolantes et faisant fi de l'acceptabilité sociale, environnementale et touristique de tels projets, tout cela, pour l'essentiel, sur le dos du contribuable français. Alors que les contraintes d'urbanisme ne cessent de limiter les prérogatives des communes, il semble qu'en l'espèce tout soit possible, en dehors de toute règle ! À écouter le Président de la République attester lui-même que « le consensus autour de l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays ». Mais sachant que l'on ne donne qu'un avis consultatif aux maires, même si le Sénat propose d'y remédier, et qu'on ignore les citoyens, comment s'étonner de la perte de confiance dans la cohérence de l'action publique territoriale ?

Cette commune, située au pied du Plomb du Cantal, à quelques pas de la vallée de Brezons, la plus belle vallée glaciaire d'Europe selon Haroun Tazieff, se voit imposer l'implantation d'un mât de mesure sans que les expressions municipales et locales aient été entendues. une durée comprise entre un et quatre ans. Comment la commune et son intercommunalité peuvent-elles, dans ces conditions, faire avancer sereinement leurs projets ? Comment les habitants peuvent-ils vendre leurs maisons avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête ? Comment accueillir de nouvelles populations demandeuses de nos espaces et de nos paysages ?

la consommation d'électricité va augmenter dans les années à venir ; il sera donc nécessaire de mettre en service de nouvelles installations de production d'électricité décarbonée. Il est donc en effet crucial d'augmenter nos capacités de production d'énergie renouvelable électrique, mais dans la concertation et en favorisant l'acceptabilité des projets- je vous rejoins. L'éolien terrestre est une des énergies renouvelables les plus compétitives ; il contribue significativement à notre sécurité d'approvisionnement, enjeu clé. En 2019, le parc éolien français a permis d'éviter l'émission de 15 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de la circulation annuelle de près de 8 millions de véhicules. Ces éoliennes sont soumises à une réglementation stricte : elles doivent obtenir une autorisation environnementale préfectorale préalablement à leur implantation, afin de démontrer que les dangers et les inconvénients du projet pour les populations, la biodiversité et les paysages peuvent être prévenus. En particulier, tout développeur éolien fournit une analyse de l'impact paysager du projet- vous m'interpellez sur ce point également -, qui est incluse dans la demande d'autorisation. Enfin, les projets éoliens doivent respecter les dispositions des documents d'urbanisme, en particulier celles du plan local d'urbanisme, le PLU, quand il existe. Pour mieux associer les riverains et les collectivités, il est surtout important de mieux planifier le développement de l'éolien en prenant en compte les spécificités locales. Le Gouvernement a

d'une procédure d'enquête très musclée et d'un interrogatoire qui n'avait rien à voir avec les faits, tout cela sur simple dénonciation, sans preuve formelle et sans que l'intéressée soit avertie au moment des faits. Autre

ce qui est des procédures judiciaires, les inspecteurs de l'environnement de l'OFB, comme leurs homologues des services déconcentrés de l'État, agissent sous l'autorité des parquets. Ils instruisent sur saisine, en toute objectivité, comme le font d'autres officiers de police judiciaire.

hiérarchiser les actions de contrôle en fonction des enjeux propres à chaque département et d'assurer la bonne coordination entre services. La bonne connaissance des milieux et des acteurs permet aux agents de l'OFB, qui sont souvent des personnalités locales, de tisser ce dialogue, cette concertation, ce partage, sur les enjeux de préservation de la biodiversité ; ainsi peut-on faire cesser les infractions et remettre en état les milieux.

Il ressort des conclusions du rapport analysant l'accident, d'une part, que l'entreprise Tereos n'aurait pas respecté la réglementation, l'entretien des bassins et digues n'étant pas satisfaisant, et, d'autre part, que la prise de conscience par les services de l'État de la gravité de la pollution aurait été trop tardive. En effet, les services compétents pour la qualité de l'eau n'ont pas été associés dès le début à la gestion de l'accident. Aucune coordination des services de l'État n'a ensuite été mise en place pour organiser le suivi de la pollution. De plus, des acteurs qui auraient pu contribuer à la surveillance du milieu aquatique et à la gestion de ces conséquences n'ont été ni informés ni associés. Enfin, les autorités compétentes en Belgique n'ont pas été prévenues à temps. Ces manquements successifs de l'entreprise et des services de l'État posent question.

Un protocole définissant plus précisément le rôle des différents services de l'État en cas de pollution touchant les milieux aquatiques et impliquant pleinement l'Office français de la biodiversité (OFB) est en cours de finalisation. Un comité de pilotage relatif à la restauration écologique de l'Escaut a été mis en place- il s'est déjà réuni trois fois -et associe toutes les parties prenantes, dont les riverains. Par ailleurs, l'inspection des installations classées a inspecté chaque site agro-industriel des Hauts-de-France comportant d'importants bassins de lagunage dès 2020. La remise en eau des bassins, elle, n'a été autorisée qu'après la réalisation d'études et de travaux. Concernant la question de la responsabilité pénale, une procédure judiciaire est en cours, qui devra déterminer les causes de l'accident, ainsi que les manquements imputables à l'exploitant. En parallèle, le préfet va engager la procédure en responsabilité environnementale de Tereos. Dans ce cadre, Tereos a admis sa responsabilité sur le linéaire français. Cette procédure permettra de prescrire à l'exploitant les mesures de réparations environnementales adaptées après qualification des dommages causés par la pollution. Après arrêté préfectoral et sur proposition d'un groupe d'experts intégrant les parties prenantes, sera présentée prochainement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) du Nord une prescription de restauration des zones d'habitat propices à la reproduction piscicole sur plusieurs secteurs de l'Escaut. Enfin, le ministère a mis en place un dispositif de vigilance renforcée pour les sites faisant l'objet d'incidents réguliers ou de non-conformité. Tereos en fera bien évidemment partie. La parole

Depuis plusieurs années, les organismes publics, notamment ceux chargés de la gestion environnementale et de la gestion de l'eau, exercent une pression forte sur les propriétaires de moulins à eau et les communes possédant des moulins sur leur territoire. Au nom de la continuité écologique, il leur est en particulier demandé de procéder à des travaux importants, dont l'arasement du vannage des moulins à eau, c'est-à-dire l'abaissement de la crête de l'ouvrage. Ces ouvrages sont, en effet, jugés responsables d'altérer le fonctionnement écologique et la biodiversité des rivières et cours d'eau. Outre le fait que la prise en charge de ces travaux est hors de portée financière pour la plupart des propriétaires, il n'est pas établi que ces vannages soient à l'origine de la dégradation de la faune et de la flore constatée depuis quelques décennies dans nos rivières. Au contraire, beaucoup d'acteurs locaux considèrent que la destruction des vannages des moulins entraîne des conséquences néfastes et irréversibles sur l'hydraulique des rivières. Elle s'accompagnera, selon eux, d'une réelle Parmi ces conséquences, on relève l'accélération du courant, la modification des berges, l'aggravation des crues, ainsi que des étiages très importants en cas de manque de pluie. Les vannages permettent, en effet, de stocker l'eau dans des zones humides ou inondables afin de prévenir les inondations en aval. aval. Il semble donc indispensable de repenser cette politique d'arasement et d'opérer des concertations locales les plus larges possible avant d'imposer des travaux coûteux dont l'intérêt semble discutable.

est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Janssens, vous m'interrogez sur les opérations réalisées sur les vannages des moulins, notamment sur les enlèvements de vannage dans le cadre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. C'est un débat que nous avons eu très largement ici même, ainsi

ont amené les parlementaires à adopter une disposition qui exclut l'effacement des seuils comme solution de restauration des continuités écologiques, à la suite de quelques dossiers territoriaux litigieux qu'il aurait fallu réexaminer de plus près. En tout état de cause, le réchauffement des eaux, la concentration des sédiments et des pollutions, le remplacement d'espèces d'eau courante par des espèces plus banales, adaptées aux eaux stagnantes, la disparition d'habitats diversifiés liée à la variation des niveaux d'eau d'une rivière courante et dynamique,

En effet, l'énergie de l'eau n'est plus dissipée par le transport des sédiments et des cailloux. Retirer des vannages obsolètes lorsque le propriétaire ne souhaite plus plus investir dans leur préparation, leur gestion et leur entretien au quotidien était une option avantageuse à la fois pour l'écologie et pour le propriétaire. C'est d'ailleurs un point sur lequel la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat,

trouver des solutions d'entretien et de gestion performantes du point de vue environnemental pour assurer cet objectif de restauration des continuités, même si ces dernières sont plus coûteuses. Je demeure évidemment à l'écoute des différents porteurs de projet. J'ai d'ailleurs proposé que nous nous retrouvions

de la transition écologique. Madame la secrétaire d'État, j'ai été alertée du problème engendré par une demande de plan de gestion qui menace gravement le mode de gestion appliqué depuis des siècles dans la forêt usagère de 3 800 hectares

d'un statut unique en Europe, qui élève les arbres au rang de bien commun mis à la disposition de la population locale. Leur prééminence sur le droit forestier a été rappelée en 1983 par la Cour de cassation. Cette décision avait réaffirmé qu'est « interdite toute coupe de bois qui ne serait pas autorisée par les syndics généraux de la forêt usagère, et ce exclusivement dans le cadre de l'exercice des droits d'usage

et mettrait fin à ce mode de gestion vertueux et respectueux de l'environnement, en place depuis plus de cinq cents ans. Depuis des siècles, l'absence d'exploitation sylvicole industrielle préserve l'intégrité génétique des pins

transactions », datant du XV siècle. Ce site classé constitue un espace naturel littoral très sensible et fragile, qui se caractérise par la diversité de la végétation. Ce mode de gestion sylvicole très original, fondé sur ces droits d'usages ancestraux, constitue un élément du patrimoine culturel local. Il explique aussi, d'ailleurs, la richesse écologique de cette forêt, qui mérite d'être préservée. Au titre du site classé, l'instruction de la demande d'approbation de ce plan de gestion auquel vous faites référence a fait l'objet d'avis favorable par les services de l'État et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. C'est dans ce cadre que l'accord du ministère pour l'autorisation de ce plan de gestion au titre du site classé a été sollicité,

Il est primordial que la situation s'apaise et que chacun puisse exercer ses droits et usages sur cette zone. Nous avons donc choisi de surseoir à toute décision sur ce plan de gestion et de diligenter une mission d'inspection, qui formulera des propositions pour concilier la protection de ce patrimoine forestier naturel et culturel original avec les enjeux de résilience des peuplements forestiers, dans un contexte de changement climatique et de maîtrise des risques incendie. Nous nous intéresserons également aux modalités de gouvernance et de dialogue à adopter dans ce contexte très spécifique de la forêt usagère. Nous serons donc tout à fait mobilisés et pleinement attachés au respect de ces enjeux.

Merci,